En application de l'article 46 , alinéa 2, du règlement du Sénat, et afin de faciliter l'organisation de nos débats, la commission des finances demande l'examen séparé des amendements n

Monsieur le ministre, vous l'avez bien compris, puisque vous orchestrez une campagne d'information- petite campagne, car vous connaissez les limites de vos propositions -pour afficher ce que vous présentez comme une formidable baisse de l'impôt, qui serait l'une des réponses importantes à la crise sociale qui secoue notre pays depuis plus d'un an. Tout d'abord, vous éludez totalement la question de la TVA- nous en avons débattu hier -, impôt injuste et massif, et vous ne criez pas sur les toits que vous réduisez, encore une fois, l'impôt sur les sociétés.

en revanche masquer cette évolution réelle et constatée : au terme des trois premiers budgets de votre gouvernement, un Français au deuxième décile- terme très apprécié à Bercy

en outre que notre proposition serait moins coûteuse pour les finances publiques que celle du Gouvernement : monsieur le ministre, nous pouvons donc collectivement faire mieux et moins cher ! Je ne doute pas que vous nous souteniez dans cette démarche. La parole est à M. Julien Bargeton, l'article. Nous abordons un article très important, qui baisse l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros pour les classes moyennes. Comme pour ce qui est de la taxe d'habitation, je cherche toujours un amendement de suppression de l'article

C'est une correction par rapport à ce qui avait été fait sous le précédent quinquennat, notamment la refiscalisation des heures supplémentaires. Je ne peux pas ne pas insister sur le gain qu'apporte le présent

Par votre promotion de la baisse de cet impôt, monsieur le ministre, vous tentez encore, un an après, de dévoyer les exigences sociales. La colère contre la taxation des carburants n'était pas l'expression d'un ras-le-bol contre l'impôt sur le revenu. Si exigence il y a concernant cet impôt, c'est celle d'une meilleure progressivité et d'une participation efficace des habitants les plus riches de notre pays à la solidarité nationale. Nous connaissons le rêve libéral : celui d'une société sans impôt, d'une société sans solidarité nationale, d'une société où règne la loi de la jungle Les promesses sont là : vous baissez un peu les impôts pour les plus pauvres de ceux qui en paient, mais, en parallèle, vous cassez les services publics ; l'exemple de l'accès aux soins est celui qui frappe le plus en ce moment. Dans le même temps, vous vous attaquez aux retraites en répondant avec empressement aux désirs du sacro-saint marché. Votre effet d'annonce d'une petite baisse d'impôt pèse bien peu face aux conséquences dévastatrices pour le pouvoir d'achat de la réforme annoncée des retraites, qui suscite décidément de plus en plus d'inquiétudes. nous, nous proposons de taxer à 60 % les plus hauts revenus, ce qui concerne environ 0,4 % des contribuables. Est-ce excessif ? Ces gens pour qui le revenu fiscal ne reflète qu'une part souvent minime de leurs revenus fréquemment défiscalisés, ne peuvent-ils mettre la main à la poche pour aider à faire face aux justes exigences du peuple ? Nous demandons justice, et rien que cela : justice, pour permettre à l'immense majorité de la population de vivre dignement ; justice, pour permettre à notre jeunesse d'espérer.

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose, à son article 13 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune

que je comprends, mais nous pensons que la baisse d'impôt décidée pour les ménages comme pour les entreprises participe au fait que notre croissance reste importante et permet des rentrées fiscales par un effet positif, notamment les rentrées de TVA.

crée un vrai problème de redistribution. On peut tenir de grands discours, mais la redistribution vers les bas revenus est faite par les prestations sociales, car l'impôt sur le revenu finance les politiques d'État qui ne sont pas redistributives. C'est bien la sécurité sociale qui est la partie redistributive.

incitative en faveur de la démographie. Comme Jérôme Bascher l'a dit à l'instant, la redistribution s'effectue par les prestations sociales, mais l'impôt sur le revenu a une vocation incitative pour l'ensemble de la population.

Voilà le fameux grand écart dans ce pays, cette fracture sociale que beaucoup ont décrite et condamnée, mais n'ont pas combattue en son temps ! Voilà la réalité ! De qui parle-t-on quand on veut faire payer les très hauts revenus ? J'ai sous les yeux le barème avec les revenus fiscaux par référence et par tranche.

Nous avions adopté un amendement visant à permettre aux élus des communes de moins de 3 500 habitants de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu 1,25 fois le montant de l'indemnité versée aux maires de communes de moins de 1 000 habitants à la condition du renoncement au remboursement des frais de transport et de séjour. En réalité, une telle condition est source de difficultés pour les élus concernés, qui ne peuvent pas savoir avant la fin de l'année s'il vaut mieux demander le remboursement de ces frais ou

M. Jean-François Longeot. Jusqu'à l'instauration en 2017 du prélèvement à la source, les élus locaux disposaient d'un système d'imposition de leurs indemnités qui tenait compte du caractère singulier de la mission qu'ils assurent sur l'ensemble du territoire de la République au service de leurs concitoyens. Ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire. Elles sont la contrepartie des sujétions imposées par leurs fonctions et de l'absence de remboursement d'une grande partie des frais qu'ils engagent. La réalité est que certains élus de petites communes sont parfois contraints d'avancer de l'argent ou en sont même « de leur poche ». Rappelons-le, lors de la fixation des critères déterminant le montant du régime indemnitaire des élus locaux dans la loi de 1992, l'esprit du législateur était clairement précisé dans la circulaire du 15 avril 1992 : l'indemnité de fonction allouée aux élus locaux « ne présente le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque Lors de l'instauration de la retenue à la source, ce dispositif légitime a été réduit et limité aux seules communes de 500 habitants et moins, ce qui aboutit à soumettre l'ensemble de la cohorte des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants à une fiscalisation de leur indemnité, au titre de la catégorie des traitements et salaires, alors que celle-ci est destinée à compenser des sujétions et des frais engagés, sans remboursement de la part de la collectivité, qui ne dispose pas des moyens de le faire. Le présent amendement vise à affranchir de l'impôt les indemnités des maires des communes situées dans les strates inférieures à 3 500 habitants, afin de redonner confiance aux maires des petites communes. Il s'inscrit dans la philosophie du projet de loi Engagement et proximité, qui tend à revaloriser l'engagement et la

d'autant plus que ces élus sont souvent amenés à financer de leur poche certaines dépenses utiles à la collectivité. Le projet de loi Engagement et proximité, tel qu'adopté par le Sénat, a apporté en partie des réponses, en revalorisant le régime indemnitaire. Toutefois, la décision revient aux conseils municipaux.

avec l'accord du Gouvernement. Sans réduire plus l'avantage fiscal qui existe pour les maires des communes de moins de 3 500 habitants, il est suggéré d'introduire un avantage un peu supérieur pour les maires des petites communes de moins de 500 habitants, à hauteur d'environ 1 800 euros.

il existe à l'hôpital un malaise persistant, un manque de personnel et des difficultés de gestion considérables.

total. Monsieur le rapporteur général,

il faudra recruter pour avoir un personnel stable et plus nombreux dans les hôpitaux. En attendant, plutôt que d'avoir des personnels de l'extérieur qui viennent faire quelques heures,

la seule solution, mais nous sommes à la recherche de solutions. Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE votera, je le répète, l'amendement de M. Karoutchi.

Les frais d'abonnement aux transports en commun engagés en vue d'effectuer des déplacements professionnels sont déductibles dans les conditions de droit commun, sous réserve, d'une part, d'être effectivement supportés par le salarié- c'est-à-dire la quote-part évoquée par le rapporteur -et, d'autre part, de ne pas être couverts par ailleurs par des allocations spéciales.

Il s'agit uniquement d'une limite au-delà de laquelle le salarié doit, pour pouvoir déduire les frais engagés, justifier de circonstances particulières d'éloignement, expliquant l'éloignement entre ces deux points. Il peut s'agir notamment de circonstances liées à l'emploi,

Il vise à créer une réduction d'impôt sur le revenu pour les versements effectués au titre de souscription en numéraire réalisés au profit d'une société coopérative ouvrière de production

Régie par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, cette formation permet notamment de généraliser l'enseignement des gestes qui sauvent. Afin d'inciter le plus grand nombre de nos concitoyens à la suivre, il est proposé d'instaurer une incitation fiscale. Il s'agit de toute évidence, mes chers collègues, d'une mesure d'intérêt général.

Pour les personnes qui bénéficient tous les ans de réductions d'impôt, cela aboutit à leur prélever un montant d'impôt artificiellement surévalué, avec un remboursement en août de l'année suivante. Pour tempérer cet effort de trésorerie du contribuable, la loi prévoit que certaines réductions d'impôt donnent lieu au versement d'un acompte en janvier. Mais toutes les réductions ne sont pas concernées, alors même que cela peut représenter des montants importants. Ainsi, un contribuable qui efface la totalité ou quasi-totalité de son impôt avec une réduction se voit quand même prélever d'un impôt théorique qui n'est pas dû, et il doit attendre plus d'un an avant d'être remboursé. Les contribuables peuvent moduler à la baisse le montant des prélèvements, mais cela n'est possible qu'en cas de diminution des revenus. Cet amendement tend à offrir la possibilité aux contribuables de moduler à la baisse leur taux de prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu en tenant compte des réductions ou crédits d'impôt auxquels leurs dépenses ouvrent droit. Quel est l'avis de la

pour la fonction publique territoriale. Les autres amendements présentés posent deux difficultés. Tout d'abord, concernant les agents expatriés de la fonction publique hospitalière, ils restent domiciliés fiscalement en France, s'ils répondent aux conditions de droit commun- avoir en France son foyer, c'est-à-dire le centre de ses intérêts familiaux ou économiques. Ce sont des règles qui s'appliquent à tous les expatriés.

l'article 2 . Cet article qui a été ajouté à l'Assemblée nationale crée une niche supplémentaire, car il prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. publique. L'ensemble des revenus et des gains, fussent-ils seulement ponctuels, honorifiques ou de remplacement, devraient être fiscalisés au titre de l'imposition des revenus, sans dérogation ou niche injustifiée. L'élargissement de l'assiette imposable est le préalable à une simplification et à une baisse des taux de notre système de prélèvements. Quel est l'avis de la commission ?

compensatoire de rupture conventionnelle sera calculée dans le secteur public comme dans le secteur privé, avec le même type de référence à l'ancienneté pour ce qui concerne l'indemnité minimale. Dans le secteur privé, je le répète, l'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée d'impôt et de cotisations sociales ; au-delà de ce qu'a déjà indiqué M. le rapporteur général et que je partage, il paraît juste que les agents du secteur public qui ont recours

: La parole est à M. Ronan Le Gleut. Cet amendement vise à revenir sur l'article 119 A de la loi de finances pour 2019 qui soumet à un prélèvement à la source de 12,8 % les dividendes d'origine française perçus par nos compatriotes établis hors de France. Ce prélèvement est ressenti comme une injustice par ces contribuables qui sont désormais obligés de prouver que leurs investissements ne relèvent pas de l'évasion fiscale. Cet amendement tend donc à l'abrogation de cet article.

que le gain fiscal lié à la réforme n'a été que très partiellement réinvesti dans les entreprises françaises compte tenu notamment des déperditions dans la consommation courante et des investissements réalisés dans le reste du monde. Plus généralement, les études empiriques les plus récentes suggèrent que l'allégement de la fiscalité au niveau de l'épargnant-actionnaire n'exerce pas d'effet sur l'investissement. Par ailleurs, la baisse du nombre de départs de redevables de l'ISF observée en 2017- une diminution de 256 -, à supposer qu'elle soit directement liée à la mise en place de l'IFI, ce qui reste à prouver, représente moins de 0,1 % du total des redevables

60 ans, suggère que la plupart n'étaient pas sur le point de démarrer un nouveau projet d'entreprise. Au total, il apparaît ainsi que la suppression de l'ISF qui constituait une forme d'imposition populaire au rendement particulièrement dynamique répondait avant tout à des motifs En outre, sur le plan de l'équité, le choix du Gouvernement de ne taxer désormais que la seule richesse immobilière a accentué les défauts de l'ISF. La réforme a conduit à exonérer totalement de très hauts patrimoines financiers- 18 % des redevables de la dernière tranche de l'ISF ne payent pas l'IFI alors même que de nombreux redevables de l'ISF restent assujettis à l'IFI sans pour autant disposer de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés- 20 % des redevables de l'IFI ont un revenu fiscal de référence inférieur à 62 000 euros.

sur notre opiniâtreté à revenir sur certains sujets ... Je ne sais pas si M. le rapporteur général émettra la même critique, mais il est vrai que nous revenons inlassablement

M. le président de la commission des finances a rappelé les chiffres lors d'une émission télévisée très intéressante diffusée cette semaine : en 2018, les cent plus grandes fortunes ont bénéficié d'un crédit d'impôt de 160 millions d'euros, soit une moyenne de 1,6 million d'euros par contribuable. Face à de tels chiffres, de dire qu'il était urgent et nécessaire d'abroger l'ISF ? Ces chiffres parlent, ils montrent l'ampleur d'un scandale que n'accepte pas notre peuple. Monsieur le rapporteur général, vous avez souligné, non sans un certain humour, les conséquences étonnantes et inacceptables de l'abrogation de l'ISF dans le rapport d'information que vous vous avez cosigné avec M. Éblé ; il y est écrit : « Paradoxalement, une stratégie indubitablement antiéconomique consistant à vendre un appartement aujourd'hui loué à titre professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yacht permet ainsi d'échapper à l'ISF ». Si cela s'est produit- et je crois que c'est le cas -, c'est proprement scandaleux ! L'adoption de notre amendement s'avère donc nécessaire. Quel est l'avis de la commission ?

L'idée d'imposer ce qui est improductif pour ramener de l'argent dans l'économie est séduisante- on pourrait y souscrire. Le seul problème, c'est qu'on a

Ce sujet avait animé nos débats l'an dernier, je vous propose de les relire aujourd'hui- certains comprendraient peut-être le ras-le-bol citoyen qui s'est manifesté alors, et pendant des mois. Le portrait social de la France présenté récemment par l'Insee devrait en tout état de cause vous conduire à conclure que la théorie du ruissellement dont vous vous prévalez ne marche pas.

Nous avons entendu les critiques de certains sur le dispositif passé et nous proposons de les corriger, tout en rétablissant une justice fiscale et une solidarité nationale. Les études économiques internationales montrent clairement que la très grande richesse est loin d'apporter à la société ce que l'organisation de la solidarité par la puissance publique est capable En d'autres termes, le monde sans puissance publique, sans État régulateur et sans solidarité nationale est un monde d'inégalités croissantes. Notre amendement va contre cette société d'inégalités et corrige les biais passés de l'ISF. Ensuite, je veux insister sur les recettes. de récupérer d'un coup d'un seul 5 milliards d'euros. Nous les apportons librement au budget de la Nation. Servez-vous-en pour financer ce que nos concitoyens réclament ! Un plan Hôpital d'envergure, une revalorisation des prestations familiales qui serait rendue possible par une compensation aux comptes sociaux des mesures visant

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Dans un contexte de hausse de la pauvreté en France, ce cadeau fiscal fait aux plus aisés n'a pas de justification. En l'absence d'accord sur le rétablissement d'un impôt

dans cette magnifique langue de Shakespeare pour laquelle j'ai le plus grand amour. Cette contribution permet de taxer les revenus du capital au taux unique de 30 %. Sont concernés les plus-values de cessions mobilières, les intérêts, les dividendes, les obligations et les revenus issus de l'assurance vie.

dont la composante immobilière est très faible, qui, pour cette raison, sont étrangères à toute logique d'investissement immobilier. En effet, lorsque les actifs imposables représentent moins de 5 % de la valeur de l'actif social, il est possible d'estimer que l'investissement n'a pas été réalisé en considération de l'immobilier sous-jacent, lequel, au demeurant, est soumis au risque d'exploitation.

Pour être tout à fait précis, dans le cas de terrains vagues, la doctrine fiscale prévoit une tolérance et admet que les réserves foncières acquises par une entreprise pour les besoins de son développement futur- seulement ceux-là -sont exclues du champ de l'IFI pendant une période de deux ans.

Cet amendement est relatif au régime de l'IFI des immeubles à valeur patrimoniale.

à la reconnaissance de la qualité patrimoniale et historique de l'édifice par une mesure de classement ou d'inscription. Elle est conditionnée par une problématique de zonage et nous proposons, dans ce cadre, de considérer les zones rurales au sens de l'Insee. Elle est conditionnée, à l'affectation du bâtiment à une activité de nature économique, qu'elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou à l'ouverture dudit bâtiment à la visite, ce qui, évidemment, participe de l'économie touristique de proximité. pensons qu'il y aurait là un intéressant dispositif de soutien au patrimoine monumental dans nos territoires ruraux. L'amendement n° I-1008 rectifié, présenté

Enfin, les instructions qui figurent dans le (BOFiP) sur l'estimation de ces biens classés précisent qu'il faut

une disposition votée à l'Assemblée nationale en faveur des propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale

Quel est l'avis du Gouvernement ?

: La parole est à M. Ronan Le Gleut. Cet amendement a pour objet de prévoir que l'effectivité de l'exercice de la fonction de direction d'un redevable doit être appréciée en tenant compte de sa présence régulière aux réunions des organes décisionnels de la société et de sa participation active aux débats et aux votes au sein desdits organes. Cette précision permettra de ne plus lier l'exonération à la seule qualité attachée aux fonctions, mais de la subordonner à une présence active à cet organe de direction, et, par voie de conséquence, de clarifier pour les redevables et sécuriser pour l'administration la notion d'effectivité, lorsque la fonction est exercée au sein d'organes de direction.

coupes, prélèvements, cueillette, d'altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives Oiseaux et Habitats ; ils sont également susceptibles de faire l'objet d'arrêtés de protection de biotopes, et plus largement, d'arrêtés portant protection des habitats naturels. Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et leurs propriétaires n'en tirent aucun revenu. Il n'est pas nécessaire d'associer au bénéfice de l'exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la

La parole est à M. Yvon Collin, pour une mise au point au sujet d'un vote. Mme Maryse Carrère et MM. Jean-Pierre Corbisez, Éric Gold, Éric Jeansannetas, Olivier Léonhardt et Jean-Yves Roux ont été notés comme s'abstenant, alors qu'ils souhaitaient voter pour.